qu'un collègue me demande, quand j'interviens, de rappeler qui je suis et d'où je viens. C'était d'autant plus gênant que je l'avais fait au cours de mon intervention ... Je veux simplement rappeler que Saint-Barthélemy

comme vous tous, et, comme tous les Français, j'ai le droit de participer, de même que les citoyens de mon île, à toutes les élections, quelles qu'elles soient, dès lors que celles-ci concernent les Français. Nous avons choisi le statut de PTOM, et nous ne sommes pas les seuls ; Saint-Pierre-et-Miquelon,

selon Légifrance, 484 textes législatifs ou réglementaires. D'ailleurs, jusqu'en 2003, l'article 4 de la loi de 1977 était rédigé ainsi : « Le territoire de la République forme une circonscription unique.

La République, c'est une idée. Les circonscriptions, ce sont des territoires. On ne peut pas diviser des idées

indispensable que les Français vivant en dehors de ce territoire puissent être représentés dans le cadre d'une circonscription spécifique ou d'une section. Encore une fois- j'ai eu l'occasion de le dire cet après-midi -, il paraît évident que les Français de l'étranger méritent d'être associés à cette construction européenne. Certes, j'ai entendu l'un de mes collègues le dire, on peut, depuis Maastricht, voter depuis l'étranger. Effectivement, l'article 8 du traité de Maastricht a permis aux Français établis hors de France ou aux Européens de voter

plutôt politique, puisque les Français de l'étranger avaient plutôt tendance à voter au centre droit- dès lors, autant les éliminer du processus

du territoire de la République- ou de la République, comme vous voudrez -en une circonscription unique, tout en préservant la représentation au Parlement européen des trois bassins ultramarins. La République constituerait bien une circonscription unique, mais, au sein de celle-ci, le scrutin serait organisé par sections pour refléter une réalité géographique. effet, selon moi, trop hasardeux de s'appuyer sur la notion de position éligible sur une liste pour assurer la présence des outre-mer au Parlement européen. Il me semble normal que la République assure et assume un reflet fidèle de son éclatement géographique sur les trois océans. Je me permets de le rappeler, cette géographie n'est pas sans incidence sur la production normative. Aujourd'hui, pour l'Union européenne, nos outre-mer sont des microproblématiques qu'elle a tendance à ne pas traiter

la représentation qu'obtiendraient les Français de l'étranger, si on les séparait du reste du corps électoral, serait minime. Vous le savez,

de la communauté nationale, dans ses composantes les plus variées, y compris celles qui ont des intérêts géographiques spécifiques ou des intérêts minoritaires de toute sorte. Nous avons d'ailleurs des collègues représentants de l'outre-mer nous affirmer qu'ils comptaient sur l'ensemble de la représentation parlementaire pour défendre les intérêts de ces territoires, et l'on pourrait dire la même chose vis-à-vis des Français établis hors de France. Il me semble donc vraiment

peuvent voter soit dans les bureaux de vote de leur poste consulaire, soit dans leur commune d'inscription en France, s'ils en expriment le choix avant le scrutin. En outre, les Français résidant dans un autre État membre de l'Union européenne et dans lequel ils ont été admis à voter peuvent voter dans leur pays de résidence pour les candidats de ce pays. Pour toutes ces raisons, je vous demande de bien

Il y a trois élus- un par bassin -, qui ont montré à quel point leur présence en Europe était nécessaire. Ils ont même été, pour certains d'entre eux- renseignez-vous -, récompensés pour la qualité de leur travail et leur défense des intérêts des outre-mer et de la France-

Quant au Conseil économique, social et environnemental, il diminuera de moitié, il y aura une disparition. Pour l'outre-mer, c'est la dilution, comme une pincée de sucre dans un grand verre d'eau

sans pour autant être à distance ni en marge de la République ! Comme si avoir des représentants élus par nos propres électeurs nous mettait en dissidence ou en marge de la République ... Ce n'est pas vrai, c'est un déni ! Je le dis ici, le Parlement n'a pas compris l'urgence qu'il y a à faire représenter les Faire élire trois représentants, ce n'est pas simplement être en dissidence ou en marge, c'est mieux intégrer les outre-mer.

Le scrutin est ouvert.

pas opportun, elle ne le fait pas. Au minimum, cette proposition permet de bien marquer l'affiliation de listes de candidats à des partis politiques européens et permet à ceux-ci de clarifier la manière dont ils abordent le choix du candidat à la tête de la Commission européenne, qui est un enjeu majeur, le premier enjeu auquel est confronté le Parlement européen lorsqu'il est élu. Laisse-t-il le Conseil choisir le président de la Commission européenne ou, au contraire,

Une pratique s'est développée à partir d'une initiative du parti socialiste européen à laquelle, en effet, je me suis trouvé modestement associé à l'approche des élections de 2014.

ce sont des confédérations d'organisations politiques, qui ont quelques difficultés à trouver un accord entre elles -ont choisi de présenter des candidats potentiels à la présidence de la Commission européenne, européenne, pariant sur le fait que les chefs d'État ou de gouvernement se tiendraient à l'intérieur de leur éventail. Rien, évidemment, dans les traités ne le prévoit.

dans les bulletins de vote eux-mêmes, car l'amendement de Jean-Yves Leconte est satisfait pour tout le reste : si vous voulez écrire sur votre déclaration de candidature que vous faites partie du groupement européen X ou Y et que vous allez soutenir M. ou Mme Dupont à la à la présidence de la Commission, vous êtes parfaitement libre de le faire. Le sujet, au fond, c'est celui-ci : considère-t-on par dérogation au droit en vigueur- sur le bulletin ne doivent figurer que les noms propres des candidats -qu'il faille prévoir que les partis qui le souhaitent présentent le nom d'un futur candidat à la présidence de la Commission européenne ? Il a semblé à la commission des lois que, du fait de la disparité des situations à la fois entre les pays et entre les formations politiques, ce serait un facteur de déséquilibre et d'incertitude que de faire apparaître un nom propre

en laissant penser que les électeurs votent pour le candidat mentionné à la présidence de la Commission européenne, ce qui est contraire aux principes électoraux en vertu desquels les bulletins ne peuvent pas comporter d'autre nom que celui du ou des candidats ou de leur remplaçant éventuel. Ensuite, le présent amendement semble impliquer que les futurs élus se trouveront en situation de compétence liée au moment du vote, dans une logique, au fond, de mandat impératif, ce qui est contraire à l'article 27 de la Constitution. si je comprends votre volonté de donner voix au chapitre à la méthode dite des, je tiens à rappeler que les États membres, comme le rapporteur l'a dit, sont divisés sur cette question. La France souhaite que l'esprit du traité de Lisbonne soit respecté : en application de l'article 17 du traité de l'Union européenne, le Conseil européen doit tenir compte des résultats des élections au Parlement européen afin de procéder à la désignation du président de la Commission européenne. Il appartient donc non pas aux listes de candidats, mais au Conseil européen de proposer au Parlement européen un candidat à la fonction de président de la Commission européenne. Pour toutes ces raisons, je le répète, nous sommes défavorables

ils peuvent peser. Par la suite, les candidats s'inscrivent dans des groupes au Parlement européen, et c'est dans ces groupes que la vie politique européenne et les choix se font. On ne peut donc pas les nier au moment des élections européennes. Enfin,

en 2014, grâce en particulier au parti socialiste et avec les autres partis socialistes européens, à l'émergence d'un peu plus de démocratie grâce au principe des, opère,

nous étions d'accord entre la droite et la gauche, de pousser cette avancée démocratique, de faire en sorte que le candidat du PPE, M. Juncker, devienne président de la Commission européenne. Il faut continuer dans cette voie pour renforcer le contrôle démocratique sur la construction européenne et singulièrement sur la Commission européenne.

Par cet amendement, nous souhaitons donner un droit de regard au CSA sur les consultations citoyennes. L'article 16 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication prévoit que le CSA adresse aux éditeurs de services publics comme privés des recommandations pendant les campagnes électorales. Le CSA utilise pleinement sa compétence, et ses recommandations, très étayées, sont rendues publiques, bien que la loi ne prévoie pas une telle publicité. Le Président Le Président Macron semble avoir convaincu ses partenaires européens d'organiser des consultations citoyennes sur l'avenir de l'Europe. Bien que les contours de ce type de consultations restent pour l'heure encore flous, il nous semble important de prévoir que le CSA puisse réguler la communication des différents partis politiques sur les ondes pendant ces périodes. Le Conseil a tendance à interpréter ses pouvoirs en deçà des campagnes électorales il l'a fait en 2005, il avait également émis une recommandation à destination des services de télévision et de radio. Il nous semble néanmoins préférable

lui aussi être soumis à des règles de répartition du temps de parole pour les partis politiques et les formations qui ont quelque chose à dire, car la consultation citoyenne les concerne au premier chef.

des futures élections européennes, le Président de la République a lancé une période de consultation citoyenne à compter du 17 avril 2019 sans que soit prévue soit prévue une quelconque organisation des débats radiotélévisés. Nous avons déposé cet amendement, car nous estimons nécessaire d'assurer des règles de pluralisme dans les médias, y compris lors de cette période. Si précampagne

qui souhaitent avoir une vision sur ce que fait en ce moment l'Union européenne, sur son bilan dans un certain nombre de domaines, et ce afin de recueillir les attentes, les préférences, les revendications des citoyens.

un. À notre sentiment, si l'on donnait ce pouvoir au CSA, on ne sait pas bien sur quoi il pourrait s'appliquer. J'ajoute que la question pourrait en revanche devenir tout à fait judicieuse après une réforme constitutionnelle qui confierait au Conseil économique, social et environnemental la mission permanente d'organiser des consultations de citoyens. S'agissant de ces consultations très circonscrites de précampagne dérouleront d'avril à octobre, elles doivent être aussi pluralistes et aussi impartiales que possible, l'objectif étant d'inciter les citoyens à s'intéresser à l'Europe et à participer au vote plutôt que de les orienter vers une liste ou une autre, listes qui ne seront pas encore constituées.

de l'Union européenne ; ce n'est donc pas franco-français -ne traiteront pas particulièrement du droit électoral ni de la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen.

de vote. Je n'ai pas été convaincu, mais je veux convaincre, parce que je vois bien que les arguments n'ont pas été très travaillés ... Oh ! ... et que la commission elle-même s'interroge.

comprendre les attentes ou les rejets des citoyens européens, et ce questionnaire sera élaboré par un groupe de travail au niveau de la Commission européenne, qui le dispatchera vers les vingt-sept États membres. L'organisation de ces consultations européennes

pendant lesquelles il veille au respect des équilibres. Là, ce n'est pas un objet de campagne électorale, c'est un objet de recensement ! Excusez-moi, mais le Front national, le parti communiste,

Tous les meetings qui seront labellisés dans ce cadre devront être pluralistes et ne pourront pas concerner un seul ou deux partis. Voilà l'explication

sur l'article. Autant je soutenais l'article 1, autant les articles relatifs aux temps de parole se heurtent à ma totale opposition. je suis tout à fait hostile à ce que deux candidats ou deux listes de candidats soient traités différemment et ne disposent pas des mêmes moyens de propagande. Il n'y a pas des grands candidats et des petits candidats, des grandes listes et des petites listes : il y a des candidats, et c'est l'électeur qui doit décider. Pour souligner le caractère quelque peu aberrant du système actuel,

Dans une vraie démocratie, les moyens publics doivent être attribués de manière égale entre les différents candidats. À défaut, on tombe dans des dérives que l'on a vues encore récemment en Égypte, pays pourtant soutenu par la France et considéré comme démocratique -c'est du moins ce que l'on dit lors des échanges diplomatiques entre la France et l'Égypte. au nom de la pensée politique dominante, ont insisté lourdement pour dénigrer la victoire de M. Orbán, dimanche dernier, en Hongrie, au prétexte que les moyens audiovisuels l'avaient favorisée. c'est exactement ce qui se passe actuellement en France : les petites listes auront deux minutes de temps de parole dans la propagande officielle, soit vingt fois moins que les listes les plus favorisées. C'est quand même une curieuse conception de la démocratie que de concentrer les moyens de propagande au profit de listes arbitrairement considérées comme plus sérieuses que les autres. Si le critère est celui des sondages, il n'y a alors plus qu'à supprimer les élections et se contenter de faire un sondage Quoi qu'il en soit, dans la mesure où le système favorise certaines listes, il est normal que les autres aient une compensation, d'où l'idée que la longueur de la profession de

est symbolique, mais il faut bien voir que le véritable enjeu des élections européennes, ce n'est pas un combat entre la droite et la gauche : c'est le choix entre une Europe des nations et une Europe fédérale.

D'autres, nombreux également, préfèrent voter pour une liste de leur pays de résidence dans l'Union européenne. Néanmoins, comment ne pas s'interroger sur ces taux de participation ?

Nous apprécions les efforts réels accomplis par ces derniers, qui doivent, hélas ! composer avec des budgets contraints, et donc des moyens limités. Il n'en reste pas moins qu'il est urgent d'agir compte tenu de l'importance concrète de l'Europe pour la vie quotidienne de tous les Français, où qu'ils vivent : nous le voyons bien à propos de la fiscalité, des échanges douaniers, du commerce international et de bien d'autres domaines relevant des compétences de l'Union européenne. Nous devons continuer à nous battre pour que nos compatriotes expatriés puissent s'exprimer. Quels moyens mettre en oeuvre pour favoriser la participation des Français de l'étranger à cette consultation électorale ? Le vote électronique permettrait sans nul doute à nos compatriotes installés à l'étranger de prendre part au scrutin. Ce sont des Français établis provisoirement hors de France ; il est important de les entendre et de leur donner les moyens de s'exprimer, où qu'ils soient dans le monde.

cette disposition, justifiée par la volonté de donner une plus grande légitimité au scrutin en favorisant les partis représentés à l'Assemblée nationale et au Sénat, reviendrait en fait à un certain déni de démocratie.

CRCE proposent donc la suppression pure et simple du présent article. Dans un esprit constructif, nous avons également déposé un amendement de repli visant à distribuer le temps de parole de manière à respecter véritablement le pluralisme politique français, sans favoriser injustement les grands partis. Un Parlement sans opposition pèche par manque de démocratie.

Comme le souligne M. Richard dans son rapport, ces campagnes officielles constituent une « garantie de pluralisme politique » : leur coût étant intégralement pris en charge par l'État, elles donnent l'occasion à des partis et groupements politiques de petite taille de s'exprimer sur les chaînes du service public, souvent à des heures de grande écoute. Or, alors que jusqu'à présent les règles en vigueur organisaient une égalité de temps d'antenne entre tous les partis et groupements politiques, il est ici question, comme on l'a fait en amont des élections présidentielles, en 2016, de mettre fin à cette égalité de traitement pour privilégier une approche dite « équitable ». Ainsi, la première fraction d'une heure

En revanche, la deuxième fraction de deux heures par chaîne réparties de manière égalitaire entre les partis et groupements politiques représentés à l'Assemblée nationale ou au Sénat, sera désormais distribuée par les présidents de groupe parlementaire, au prorata de leur nombre de députés ou de sénateurs.

au meilleur animateur ou à la meilleure animatrice reviendra le meilleur temps de parole ; la représentativité des listes de candidats, qui reposerait « en particulier » sur deux sous-critères, à savoir les résultats obtenus aux dernières élections européennes et aux plus récentes élections par les candidats ou « formations politiques » qui les soutiennent, d'une part, et les indications des « enquêtes d'opinion », d'autre part. On le voit bien, le caractère particulièrement subjectif et attentatoire à la démocratie de ces critères impose de modifier cette répartition du temps d'antenne ; c'est ce que nous proposerons

à adapter les modalités d'attribution des temps d'antenne lors de la campagne audiovisuelle officielle des élections européennes, en tirant les conséquences d'une décision du Conseil constitutionnel Dans son avis du 21 décembre 2017, le Conseil d'État a considéré que la mise à disposition des listes de candidats des antennes du service public de la communication audiovisuelle constitue un mode de propagande qui n'est désormais ni le plus moderne ni le plus influent dans la campagne électorale. est donc opportun de s'interroger quant au maintien de ces communications audiovisuelles. La suppression de l'envoi de la propagande officielle -circulaires et bulletins de vote -est systématiquement proposée depuis quatre ans lors de l'examen du projet de budget. Il conviendrait prioritairement de renforcer les moyens mis à la disposition des représentants de l'État pour assurer la bonne diffusion de ces documents. Les graves manquements constatés lors des élections législatives de juin 2017 illustrent les dysfonctionnements que subit la distribution

millions d'euros ... Par cohérence, il conviendra également d'abroger l'article L. 167-1 du code électoral applicable aux élections législatives, lequel a déjà été partiellement censuré par la décision du Conseil constitutionnel précitée.

Il n'est pas démocratique de décider à l'avance que tel ou tel courant d'opinion a plus de chances de l'emporter qu'un autre et de lui accorder, sous ce prétexte, des moyens considérables, lui donnant parfois un avantage décisif.

est d'autant plus vrai que l'effectif des groupes parlementaires n'est absolument pas représentatif de l'audience électorale. Par exemple, en 2012, au premier tour de l'élection présidentielle, le Front national a obtenu 6 421 426

élections législatives de 2017, des distorsions du même type ont été observées. Compte tenu du scrutin majoritaire et des tractations politiciennes qu'il permet, il est donc évident qu'une répartition du temps de parole au prorata des groupes politiques du Parlement n'est pas du tout représentative de l'audience des divers courants d'opinion.

qui est la matrice de l'article 2 de ce projet de loi, le Conseil constitutionnel a censuré le dispositif applicable aux élections législatives, au motif qu'il permettait une répartition du temps de parole « hors de proportion » avec l'état réel des forces politiques du pays, bouleversé par la percée du mouvement En Marche ! Cette expression a été intégrée à la rédaction de l'article 2 afin d'en garantir la constitutionnalité. En adoptant une approche globale, nous considérons toutefois que ces précautions ne sont pas suffisantes, dès lors que la part minimale de temps de parole attribuée à chaque liste est considérablement réduite dans le cas des élections européennes.

texte. Mais, en fonction des calculs établis par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dont les modalités restent à expliciter, les temps de parole vont considérablement varier d'une liste à l'autre. Cette situation pourrait alimenter le sentiment de censure chez une partie de nos concitoyens.

Je comprends l'argument invoqué par M. le rapporteur, qui craint une multiplication des listes, en l'absence de parrainages. Toutefois, à mon sens, l'allongement des débats est préférable à une censure trop rigide des nouvelles formations politiques. Plusieurs d'entre nous considèrent que les débats relatifs à l'Union européenne occupent une place trop marginale au regard du rôle désormais important que joue le Parlement européen dans l'équilibre institutionnel bruxellois. L'allongement de la durée minimale de temps de parole pourrait permettre aux citoyens de mieux juger de la qualité d'un programme et de l'aptitude au débat démocratique d'un candidat.

d'émission du service public de la communication audiovisuelle qui garantit l'expression pluraliste des opinions en France. Comme nous l'énoncions en défendant notre amendement de suppression de l'article 2, la nouvelle répartition du temps d'antenne proposée par le Gouvernement, qui s'appuie sur un principe d'équité, ne nous paraît

Rien ne justifie que les formations majoritaires soient favorisées- elles le sont déjà tout au long de l'année ! -, au détriment du nécessaire renouvellement du paysage politique français. Il nous faut au contraire encourager la diversité des listes électorales lors des élections européennes et ne pas nuire à la bonne information des électeurs sur les partis ou groupements politiques souhaitant accéder au Parlement européen.

Le mécanisme du scrutin majoritaire et les tractations politiciennes lors du second tour ont pour conséquence que les résultats des élections législatives, en nombre en nombre de sièges, ne reflètent ni les résultats en nombre de suffrages obtenus ni l'audience réelle des courants d'opinion exprimés lors du scrutin. La constitution des groupes politiques aggrave encore ce constat. Prendre en compte ces derniers revient purement et simplement à rayer d'un trait de plume les partis dont les parlementaires ne sont pas assez nombreux pour constituer un groupe. Après avoir été victimes du scrutin majoritaire, ces partis sont victimes de la priorité donnée aux groupes, ce qui constitue une caricature de démocratie.

M. David Assouline. Nous disposons désormais d'une jurisprudence constitutionnelle permettant de clarifier la méthode que le législateur doit employer pour répartir le temps de parole durant les campagnes audiovisuelles officielles précédant les élections. Le Conseil constitutionnel a estimé, dans sa décision du 31 mai 2017, que le législateur ne peut pas octroyer aux partis et groupements politiques non représentés à l'Assemblée nationale un temps d'antenne manifestement hors de proportion avec leur représentativité ». Cela méconnaîtrait l'obligation constitutionnelle de maintien du pluralisme et de participation équitable des partis et groupements à la vie démocratique de la Nation. Vraisemblablement, l'équilibre entre les deuxième et troisième fractions, tel que prévu dans le projet de loi, ne répond pas à cet objectif, dans la mesure où deux heures sont octroyées aux grands partis représentés nationalement, à charge pour le CSA de répartir l'heure restante entre tous les autres candidats.

La solution qu'il propose, et qui a été adoptée par la commission des lois, constitue une légère avancée, puisqu'elle permettra au CSA de disposer de plus de souplesse et de davantage de temps de parole à distribuer pour

à chaque parlementaire et à supprimer les références aux groupes parlementaires, afin de garantir un plus grand pluralisme, puisque les parlementaires n'appartenant pas à un groupe seraient, eux aussi, pris en considération, et une meilleure représentativité, puisque puisque tous les parlementaires bénéficieront du même poids dans le calcul de la répartition. Enfin, l'adoption de cette rédaction permettrait de faciliter l'application des dispositions faisant référence aux notions de « partis et groupement politiques » et « d'inscription et de rattachement », qui ne sont pas définies juridiquement et peuvent prêter à confusion. C'est pourquoi nous proposons de préciser par décret en Conseil d'État les conditions d'inscription et de rattachement des députés, des sénateurs et des représentants français au Parlement européen aux partis et groupements politiques. L'amendement n° 38, présenté par M. Assouline,

négociation les responsables des partis non représentés nationalement ; elle interdit le soutien à plusieurs listes qui pourraient être issues d'un même groupe parlementaire « national » ; elle favorise ainsi, de fait, l'expression des grands partis ; enfin, la répartition étant effectuée loin des instances européennes, elle ne constitue pas la solution la mieux à même de garantir la transparence. Pour ces raisons, la solution retenue par le texte me semble être de nature à porter atteinte au principe constitutionnel de maintien du pluralisme au sein des médias. Notre amendement vise donc à permettre aux chefs des délégations françaises

Dans ces conditions, un groupe politique ne peut pas sérieusement prétendre qu'il est légitime qu'il soutienne simultanément plusieurs listes. Dans son avis sur le projet de loi, a d'ailleurs lui-même demandé l'application de la règle selon laquelle chaque parti ou groupement politique ne peut soutenir qu'une seule liste.

joué par les sociétés Facebook et Cambridge Analytica lors des élections américaines et du référendum sur le Brexit renforce les suspicions du public à l'encontre des nouveaux géants médiatiques. couper court à toute théorie du complot, nous souhaitons que la répartition des temps de parole lors des prochaines élections européennes se déroule dans les conditions le plus transparentes possible. Tel est l'objet du présent amendement, qui vise à ce que la répartition des temps de parole opérée par les groupes parlementaires

L'objet de cet amendement est d'inscrire cet objectif constitutionnel d'expression du pluralisme dans le dispositif de répartition du temps de parole géré par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, afin qu'il ne soit pas trop défavorable aux formations politiques non représentées au Parlement. En l'état actuel du texte, les critères de répartition sont assez flous, notamment en ce qui concerne la mention relative aux instituts de sondage. Cela pourrait renforcer la dimension de prophétie autoréalisatrice des débats ainsi organisés. Il s'agit également de ne pas assujettir le débat relatif aux élections européennes aux mêmes contingences que les campagnes des élections nationales, en cohérence avec notre volonté de promouvoir le développement de listes transnationales.

attribuées au titre des deux autres fractions, qui permettent d'aboutir à un juste équilibre. Je tiens à rappeler que, lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale, le Gouvernement a déjà accepté de porter le forfait de deux à trois minutes.

plusieurs difficultés, dès lors que la deuxième fraction serait attribuée à des partis politiques, tandis que la première et la troisième reviendraient aux listes de candidats.

Concernant l'amendement n° 4, en mettant les deux heures de la deuxième fraction à disposition des présidents de groupe, le Gouvernement a souhaité s'en remettre à la sagesse de ces derniers et à celle des groupes parlementaires. Mettre en oeuvre cette répartition est également plus simple qu'organiser un système complexe de parrainage de plusieurs centaines de parlementaires. L'avis est défavorable. qui concerne l'amendement n° 37, le dispositif que propose le Gouvernement vise à maintenir une durée plus importante de temps d'antenne pour les listes soutenues par des formations représentées au Parlement. Cette prime donnée à la représentation parlementaire existait précédemment

Pour que ce mécanisme correctif fonctionne, il ne doit pas conduire à attribuer une même durée d'émission que le mécanisme principal, fondé sur la représentation parlementaire. L'avis est défavorable.

S'agissant de la prise en compte des représentants français au Parlement européen comme déterminant de la répartition des temps d'antenne, je tiens à préciser que cela est d'ores et déjà prévu au travers de la troisième fraction.

de la troisième partie parce que ces résultats ne permettent pas de donner une image suffisamment actualisée des rapports de force politiques, les dernières élections européennes ayant eu lieu en 2014.

et des présidents de groupe à l'Assemblée nationale et au Sénat viendrait complexifier l'économie du projet. En outre, les personnes qui seront candidates aux élections européennes de 2019 ne l'étaient pas nécessairement lors du précédent scrutin européen

Au contraire, la formulation proposée à l'article 2 s'inspire directement de la décision du Conseil constitutionnel et me semble plus précise. En effet, elle indique clairement que l'objectif de la fraction de correction est d'éviter l'attribution à certaines listes

France 2, France 3, France 4, France 5, France O et Réseau France Outre-Mer pour France Télévisions ; France Inter, France Info, France Bleu, France Culture, France Musique, le Mouv'et FIP pour Radio France ; France 24, RFI et Monte Carlo Doualiya pour France Médias Monde.

de la campagne électorale en vue des élections législatives. Dans sa décision, le Conseil constitutionnel a fixé au 30 juin 2018 la date de l'abrogation de ces dispositions, afin de laisser au législateur le temps de les remplacer. Il est apparu opportun au Gouvernement d'utiliser le présent vecteur législatif pour se conformer à cette décision dans ce délai et éviter ainsi l'apparition d'un vide juridique. Or le présent projet de loi relatif à l'élection des représentants au Parlement européen ne visait initialement que la loi du 7 juillet 1977, et nullement le code électoral. Conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, il est proposé de supprimer cet article, qui est à l'évidence un cavalier législatif.

des élections législatives, moment fort du débat démocratique, n'est pas une mince affaire. C'est une question très complexe sur le plan technique et qui peut avoir de lourdes conséquences politiques. Comment

de plus précipitée puisque les prochaines élections législatives n'auront lieu qu'en 2022. Nous savons qu'elle répond à une injonction du Conseil constitutionnel en date du 30 novembre 2017. Par ailleurs, sur le contenu de cet article, beaucoup a déjà été dit à l'occasion de l'examen de l'article précédent. Je n'y reviendrai pas, sauf pour souligner à nouveau le véritable scandale démocratique que représente la substitution du principe d'équité au principe d'égalité dans les règles de calcul du temps de parole.

d'ordre subjectif. Nous préférons à celui-ci le principe d'égalité, qui prévalait auparavant. La troisième fraction du temps de parole serait répartie en fonction de la participation des partis et groupements politiques à l'animation du débat électoral.

Or nombre de chaînes d'information et d'instituts de sondage sont aux mains des puissances financières, ce qui engendre un doute sérieux sur leur objectivité. Nous vous proposons donc, au travers de cet amendement, de supprimer une disposition dangereuse pour le pluralisme. Quel est l'avis de la commission ? L'avis de la commission ? L'avis est défavorable, parce que nous ne travaillons plus sur un champ de complète liberté du Parlement. Je rappelle de temps en temps, de façon un peu fastidieuse, que le Parlement n'est pas au-dessus de l'État de droit

a énoncé un équilibre dans lequel figure en effet l'ensemble des élections antérieures. Cela signifie, par exemple, qu'une organisation politique comptant de nombreux représentants lors des élections locales

Nomination des vingt-sept membres de la mission d'information sur le développement de l'herboristerie et des plantes médicinales, des filières et métiers d'avenir.